J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi permettant d'offrir des chèques-vacances aux personnels des secteurs sanitaire et médico-social en reconnaissance de leur action durant l'épidémie de covid-19 est parvenue à l'adoption d'un texte commun. L'ordre du jour appelle la discussion en nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire

Nous aurions préféré organiser le rétablissement immédiat et total des règles de droit commun. Malheureusement, en Guyane et à Mayotte, la circulation du virus reste préoccupante. Cela explique l'article 1 de ce texte, qui proroge l'état d'urgence sanitaire dans ces deux territoires. En métropole, le virus continue de circuler. Nous avons recensé 500 nouvelles contaminations le 30 juin ; 300 foyers, ou « clusters », sont identifiés à cette date.

En effet, un travail de grande qualité avait été engagé entre les deux chambres. Un point de consensus avait été trouvé, au moins sur l'article 2, concernant les données nécessaires à la recherche et à la surveillance épidémiologique, qui a fait l'objet d'un vote conforme. Le principal désaccord avait déjà été soulevé en première lecture. Il porte sur la gestion d'un éventuel retour de l'épidémie de covid-19 au niveau local et sur les moyens donnés au Gouvernement pour l'éviter. La ligne du Gouvernement a toujours été claire : éviter tout risque de reprise de l'épidémie et être capable d'agir rapidement, sans se voir obligé de déclencher, une nouvelle fois, l'état d'urgence Ce projet de loi est la seule voie possible entre deux écueils : la sortie sèche et la prorogation. Nous savons que la réponse à la menace sanitaire doit être revue et réorganisée. C'est tout le sens de la proposition avancée par le président Bas pour tirer tous les enseignements de la crise. Lors des débats parlementaires sur la loi du 23 mars dernier, il a en effet été convenu de réviser l'ensemble du dispositif de gestion des crises sanitaires. Un débat global pour redéfinir le cadre de l'état d'urgence sanitaire interviendra ainsi avant le 1 avril 2021, comme le Sénat l'a souhaité. Mesdames, messieurs les sénateurs, ce texte tient compte d'une situation épidémique qui requiert encore une prudence individuelle et collective de chaque instant. Le risque d'une deuxième vague existe : les exemples étrangers ne manquent pas de nous appeler à la vigilance. Il nous faut des outils qui nous permettent de faire face au retour possible de clusters localisés : ce qui se passe en Allemagne nous y invite. Le Royaume-Uni durcit d'ailleurs localement le confinement : c'est le cas à Leicester, où les commerces non essentiels, qui avaient rouvert à la mi-juin, doivent à nouveau fermer. L'état d'urgence sanitaire n'a pas été mis en oeuvre par complaisance. Nous l'avons fait parce que nous n'avions pas le choix. il a été répété lors des précédents débats, le Gouvernement souhaite disposer d'outils pour éviter la propagation du virus sans avoir à rétablir l'état d'urgence sanitaire. Rappelons que celui-ci doit être justifié par une catastrophe sanitaire. En nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, nous avons souhaité rester sur cette ligne. Votre commission des lois a déposé une motion tendant à opposer la question préalable. Nos débats de ce matin seront donc probablement abrégés. Il est vrai que les désaccords constatés en commission mixte paritaire persistent. Toutefois, je me dois de rappeler que le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture tient compte de plusieurs dispositions adoptées La navette parlementaire aura pleinement joué son rôle, en permettant d'enrichir le texte et d'y apporter les corrections nécessaires. Le Gouvernement vous invite, mesdames, messieurs les sénateurs, à adopter ce texte, qui est à la fois protecteur des libertés fondamentales et adapté aux circonstances sanitaires. La parole

largement participé à l'élaboration de la loi du 23 mars dernier ; nous avons également été force de proposition en vue de l'adoption de la loi du 11 mai dernier : le Sénat a répondu présent à chacune des étapes de la lutte contre l'épidémie de covid-19, le plus grand fléau sanitaire que la France ait connu depuis près d'un siècle. Nous avons voulu, forts de cette expérience et de la qualité de notre coopération avec le Gouvernement et l'Assemblée nationale, poursuivre sur la même voie pendant la discussion du présent texte, dont le titre indique qu'il a pour objet la sortie de l'état d'urgence sanitaire. Mais nous nous sommes heurtés à une difficulté,

des principaux pouvoirs conférés par le législateur au Gouvernement pour lutter contre l'épidémie dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Nous nous sommes demandé ce que vous vouliez vraiment, monsieur le secrétaire d'État. Si vous vouliez reconduire l'état d'urgence sanitaire, rien n'était plus simple

dans sa robustesse- j'allais dire sa rusticité -, il nous a paru devoir s'imposer. C'est la raison pour laquelle nous avons adopté, en première lecture, des dispositions qui étaient strictement calibrées en fonction des besoins, ici et maintenant, exprimés par le Gouvernement. Nous estimions que, si la situation sanitaire devait de nouveau se dégrader,

à l'expiration d'un délai d'un mois, si cela lui paraissait nécessaire et justifié du point de vue de la Constitution.

pour beaucoup de nos concitoyens, l'état d'urgence sanitaire était devenu synonyme de confinement. Nous avons imaginé que le Gouvernement voulait conserver les moyens offerts par cet état d'urgence, mais sans le dire, pour ne pas traumatiser nos concitoyens, qui sortent, heureusement, de cette période de confinement. Ce n'est peut-être pas que vous vouliez le beurre et l'argent du beurre, mais vous voulez à la fois la fin de l'état d'urgence sanitaire et l'état d'urgence sanitaire. C'est du moins

une forme d'infantilisation. C'est pourquoi nous vous avons, en quelque sorte, mis au pied du mur. Nous espérions vous convaincre ; nous ne vous avons pas convaincu.

ni acrimonie, et même avec la bienveillance que le Sénat sait toujours montrer au Gouvernement. Vous le savez, le Sénat est génétiquement constructif.

l'interdiction de circuler, d'aller et de venir, la fermeture provisoire des établissements recevant du public, ce qui pose la question du droit de réunion,

Il y a là quelque chose que je comprends d'autant moins que nos collègues de l'Assemblée nationale ont souhaité supprimer

solution hybride et injustifiée qui consiste à donner au Premier ministre les pouvoirs que l'on retire en supprimant l'état d'urgence sanitaire : de fait, on ne supprime pas

il est toujours en circulation active, il fallait donner au Gouvernement les moyens de réglementer de façon ponctuelle, voire locale ; je pense notamment aux transports collectifs. Aujourd'hui, après l'échec de la commission mixte paritaire, nous en revenons au texte initial, qui n'est ni plus ni moins qu'un vrai-faux état d'urgence. L'Assemblée nationale, contrairement au Sénat, a décidé de revenir sur des interdictions, plutôt que sur des possibilités de « réglementation » comme l'avait prévu le Sénat. La prolongation, pour quatre mois, des prérogatives du Premier ministre en matière de déplacements et de règles portant sur les établissements accueillant du public ne nous choque pas outre mesure. Il n'en est pas tout à fait de même pour celles ayant trait aux rassemblements sur la voie publique : on touche là au coeur de nos libertés fondamentales. Ce qui nous dérange, c'est cette banalisation de l'exception : le passé nous a bien enseigné que, chaque fois qu'un état d'urgence a été instauré, il en est resté quelque chose dans notre droit commun. Bien trop souvent, l'exception est devenue la règle. En cas de seconde vague, un simple décret permettrait de déclarer l'état d'urgence. Si j'entends l'objectif de célérité, ces mesures vont ôter toute valeur au véritable état d'urgence. Elles viennent également affaiblir le Parlement, qui n'est même plus consulté sur un sujet d'une extrême sensibilité. On sait combien nous sommes tous attachés, dans cet hémicycle, aux libertés individuelles.

réalisables ; elles auraient garanti à la fois la protection des populations faiblement touchées, la circulation des personnes et l'activité économique.

Mes chers collègues, vous l'aurez compris, même si nous partageons sur le fond l'avis du Sénat sur ce texte profondément modifié par l'Assemblée nationale, sur lequel il n'a pas été possible

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le texte que nous examinons ce matin aurait pu être- aurait dû être, ai-je envie de dire -un texte de la commission, dans la continuité du dialogue constructif entre les deux chambres dont avait fait l'objet, précédemment, ce projet de loi. La commission des lois a toutefois fait un autre choix, en adoptant hier une motion présentée par son rapporteur. Je le déplore non pas sur le fond, puisque ce texte intègre, à nos yeux, un certain nombre de points d'équilibre et d'apports du Sénat et prend acte des principales remarques qui avaient été formulées,

La sagesse de la Haute Assemblée et la qualité des travaux de son rapporteur, M. Philippe Bas, ont en effet permis, dans un passé proche, de surmonter des points de divergence plus marqués que celui- soyons bien précis

Je souhaite rappeler les apports du Sénat, qui a justement approuvé, en première lecture, l'économie générale de ce projet de loi et le principe d'un régime transitoire de sortie de l'état d'urgence sanitaire.

et sortie sèche. Je pense à la différenciation entre le régime transitoire de l'article 1 et le régime de l'état d'urgence sanitaire, s'agissant notamment de l'encadrement des conditions de réglementation des rassemblements sur la voie publique. Je pense également aux mesures relatives à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française. D'autres dispositions avaient fait l'objet d'un compromis entre les deux assemblées : l'avancée de l'échéance du dispositif transitoire, l'article 2, relatif à la recherche et à la surveillance épidémiologique, ou encore le maintien du Conseil scientifique jusqu'au terme

Sur le principal point de divergence, à l'article 1, la rapporteure n'a pas souhaité rétablir telle quelle la disposition relative à la circulation des personnes et des véhicules. Elle s'en est tenue à une faculté d'interdiction pour les seules parties du territoire où serait constatée une circulation active du virus. Cette disposition ne permettrait en aucun cas de fonder des mesures générales et absolues

si le principe même de la navette parlementaire a un sens et ne se résume pas à une posture politicienne, il faut laisser du temps

pourquoi cette précipitation, alors que l'état d'urgence sanitaire se termine le 10 juillet ? En première lecture au Sénat, le 22 juin dernier, j'avais voté sans hésitation contre ce projet

J'avais alors dénoncé avec force le projet originel du Gouvernement, qui permettait au Premier ministre de restreindre de manière arbitraire les libertés publiques jusqu'au 30 octobre prochain, sans que le Parlement ait à se prononcer de nouveau.

supprimant la possibilité d'interdire les manifestations, mais en maintenant celle de réglementer les libertés publiques. Or chacun sait qu'une réglementation excessive, tatillonne, peut entraîner une grande restriction de droits pourtant constitutionnellement fondés. paritaire, la majorité de l'Assemblée nationale n'a pas cédé sur ce qui constitue pour elle l'essentiel. En effet, elle a réintroduit la possibilité d'interdire l'exercice de certaines libertés publiques, en premier lieu les libertés de circulation et de réunion. Certes, elle a conditionné ces nouvelles interdictions à un cadre géographique limité,

pourquoi ne pas avoir rejeté ce texte d'emblée, dès la première lecture, d'autant que nous connaissons l'aveuglement de la majorité qui soutient sans faillir Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale ? Pourquoi ce projet de loi, alors que l'article L. 3131-1 du code de la santé publique accorde des pouvoirs très larges au ministre de la santé en cas de circonstances exceptionnelles ? Comment ne pas

contestation sociale qui ne manquera pas de se développer, tant la violence de la crise s'abat sur les plus défavorisés, sur les salariés, tant l'absence de réponse aux légitimes revendications des personnels soignants choque ? Oui, il faut un état d'urgence, monsieur le secrétaire d'État, mais un état d'urgence sociale, pour accompagner les victimes sanitaires et économiques de la crise de la covid-19. L'interdiction des licenciements, l'augmentation des salaires et des minimas sociaux, le blocage des prix dans l'alimentation ou l'énergie sont des exemples de mesures à prendre dans ce cadre. Bien évidemment, vous n'évoquez pas cette urgence-là

Cela signifie retrouver progressivement nos libertés. Le projet de loi que nous examinons ce matin en nouvelle lecture a pour objet d'organiser la fin de cet état d'urgence sanitaire, en prévoyant une sorte de période de transition jusqu'à la fin du mois d'octobre prochain.

L'un des principaux points de désaccord entre le Sénat et l'Assemblée nationale concerne les menaces sanitaires et les moyens d'action du ministre chargé de la santé. La rédaction proposée par le Sénat pour l'article L. 3131-1 du code de la santé publique venait préciser les pouvoirs dudit ministre dans la lutte contre l'épidémie. Elle apportait une sécurité supplémentaire avant la révision du dispositif qui devrait intervenir au mois d'avril prochain. Nous avons été particulièrement sensibles à la restriction, parfois extrêmement importante, de nos libertés. Nous l'avions exprimé lors de la première lecture, notamment au sujet de la liberté de manifester, de la circulation des personnes et des véhicules ou encore de l'ouverture des établissements accueillant du public. Cette privation de libertés était certainement nécessaire, mais, une fois la crise passée, elle doit être levée aussi vite que possible. La gestion de l'épidémie par un retour progressif à la normale après la fin de l'état d'urgence sanitaire doit respecter un équilibre entre liberté et sécurité.

Il faut qu'ils continuent pour réduire la progression du virus sur notre territoire. Pour l'heure, ni traitement ni vaccin ne sont encore disponibles. Les précautions et la prudence doivent rester de rigueur. Nous avons aussi eu l'occasion de le dire en première lecture : la gestion de cette sortie de crise doit respecter la spécificité de chacun de nos territoires. Tous n'ont pas été touchés de la même manière ni avec la même intensité. Les mesures de gestion de l'épidémie doivent être adaptées aux différentes situations. répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'État nous semble essentielle, plus encore dans nos territoires ultramarins. Plusieurs mesures vont dans ce sens. Restons mobilisés et vigilants. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles, mais, lorsque la situation sanitaire revient progressivement à la normale, cela doit s'accompagner d'un retour progressif à la normale de notre droit.

d'adopter les dispositions proposées par le Gouvernement. Certains avaient d'ailleurs évoqué dans cet hémicycle une prorogation de l'état d'urgence sanitaire qui ne disait pas son nom En première lecture, nous avions largement débattu de l'article 1, qui conservait à l'exécutif la plupart des pouvoirs dont il disposait dans le cadre de l'état d'urgence Plusieurs de nos collègues avaient insisté sur le fait que la sortie de l'état d'urgence ne privait pas le Gouvernement de moyens juridiques suffisants pour gérer la sortie de crise. Le code de la santé publique prévoyait déjà de nombreuses dispositions de droit commun permettant à l'exécutif d'agir efficacement dans le cadre d'une épidémie. Ce sont d'ailleurs ces dispositions que le Sénat proposait d'améliorer à travers l'article 1 A, qui procédait à une réécriture bienvenue de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique. La commission des lois du Sénat avait également remodelé l'article 1. Nous avions été nombreux à nous laisser convaincre par la pertinence des aménagements présentés par le président Bas. L'objectif était simple : limiter strictement les modifications législatives à ce qui était nécessaire dans le cadre du déconfinement. Pas plus, mais pas moins, sûr la possibilité d'activer de nouveau l'état d'urgence sanitaire dans les mois qui viennent si la situation sanitaire de notre pays devait se dégrader. Ce point d'équilibre raisonnable avait convaincu une majorité des membres paritaire n'a pu aboutir. Sans surprise, la majorité de l'Assemblée nationale a presque intégralement rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture. En d'autres termes, la voix du Sénat n'a pas été entendue. Il apparaît donc logique que nous ne souhaitions pas poursuivre ce dialogue de sourds. Pour autant, je veux mettre en lumière, au nom de mon collègue calédonien Gérard Poadja, deux précisions qui ont été adoptées mardi dernier, lors de la nouvelle lecture du texte à l'Assemblée nationale, sur proposition des députés calédoniens Philippe Dunoyer et Philippe Gomès. Aux articles 3 et 4 du projet de loi, relatifs aux mesures d'adaptation du rôle du représentant de l'État en matière de gestion de l'état d'urgence sanitaire en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie, il est désormais précisé que l'exercice des prérogatives du haut-commissaire se fait « dans le strict respect de la répartition des compétences » entre l'État et la Collectivité de Nouvelle-Calédonie, d'une

est malheureux. L'entrée dans l'état d'exception représente un moment délicat de la vie institutionnelle et parlementaire, dans lequel l'unité la plus large est souhaitable ; la sortie de cet état aurait dû se faire dans des circonstances comparables. Il est vrai qu'une réelle recherche de compromis a pu avoir lieu avant et pendant la commission mixte paritaire, grâce aux efforts de notre président-rapporteur, Philippe Bas, qui, depuis le début de la crise sanitaire, incarne la démarche sénatoriale de pragmatisme sur les moyens et de fermeté sur les principes. Après ces discussions, il aurait même été possible d'atteindre un accord sur certains points. Cependant, des désaccords de fond demeuraient. Ils étaient liés à la question centrale des pouvoirs qu'il sera nécessaire de maintenir entre les mains du Gouvernement, aussi bien durant qu'après la période qui s'annonce de sortie de l'état d'urgence sanitaire. La position de notre assemblée était qu'un retour à la normale, pour être plus qu'un slogan, devait s'accompagner d'une diminution des pouvoirs spéciaux de nature coercitive accordés à l'exécutif. Cela ne nous désarme pas face au virus : nous avons toujours souligné qu'il demeurait possible de déclarer de nouveau l'état d'urgence sanitaire sur tout ou partie du territoire, si nécessaire. Rétablir l'état d'urgence sanitaire n'est pas une perspective réjouissante, évidemment, mais nous pensons que, comme les Allemands ou les Portugais, les Français sont suffisamment responsables pour accepter que soient prises les mesures qui s'imposent, et ce sans qu'il soit nécessaire de se livrer à des contorsions sémantiques et juridiques. Il faut appeler les choses par leur nom, car ne pas car ne pas le faire ne contribuerait qu'à semer le doute dans l'esprit de nos concitoyens, ce qui n'est certainement pas un gage d'adhésion aux mesures sanitaires. Telle était notre position lundi dernier, indépendamment des ajustements et adaptations qui demeuraient comme toujours envisageables en vue de la commission mixte paritaire. Cette position n'a pas changé après l'échec de cette Or le texte qui nous revient aujourd'hui de l'Assemblée nationale porte la marque d'une certaine divergence dans la compréhension de la fin de l'état d'urgence sanitaire, même s'il est vrai que quelques apports sénatoriaux y subsistent. C'est un pas dans la bonne direction, mais ce n'est pas suffisant. D'abord, l'article 1 du texte voté par les députés comprend un certain nombre de retours en arrière que nous ne pouvons accepter, en particulier le rétablissement de la possibilité d'interdire la circulation dans certaines parties du territoire. Il me semble difficile d'approuver des restrictions générales et absolues qui limiteraient la liberté d'aller et de venir, tout en proclamant le retour à la normale. Recommencer à interdire des déplacements, ce n'est pas sortir de l'état d'urgence

Une telle différence de traitement entre Français métropolitains et Français ultramarins me paraît difficilement justifiable, eu égard aux autres outils dont disposent les pouvoirs publics. Telle était déjà, par le passé, la position de notre assemblée. Enfin, les députés ont supprimé l'article 1 A, qui contenait les mesures proposées par le Sénat pour rénover l'article L. 3131-1 du code de la santé publique. Les faiblesses de la rédaction actuelle de cet article ont déjà été amplement soulignées et sont par ailleurs reconnues par le rapporteur de l'Assemblée nationale. Malgré tout, il a fait supprimer cet ajout du Sénat, en renvoyant à une date ultérieure la modernisation du régime de droit commun de gestion des crises sanitaires, alors même que nous discutons d'un texte dont l'objet est de préparer le retour au droit commun. Je suis pourtant certaine qu'un accord aurait été possible, ne serait-ce que sur un commencement d'amélioration de cet article juridiquement trop flou. Quelqu'un de plus facétieux que moi pourrait aller jusqu'à soupçonner la majorité gouvernementale de vouloir faire sien ce mot du cardinal de Retz : « On ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens.

et de revenir ainsi sur notre vote initial. Le président de notre groupe, Bruno Retailleau, l'a bien exprimé la semaine dernière : « Nous sommes parvenus à la limite de nos capacités de souplesse et nous ne pourrons accepter des dispositifs plus contraignants.

il a même fait preuve d'une approche constructive en première lecture et admis que le Gouvernement devrait conserver un certain nombre de prérogatives après le 10 juillet. Toutefois, nous constatons que les divergences que nous avons eues, en commission mixte paritaire, avec nos collègues députés se retrouvent dans le texte adopté par l'Assemblée nationale. La différence entre le régime transitoire qui entrera en vigueur le 10 juillet prochain et l'état d'urgence sanitaire demeure, en pratique, trop ténue. Bien sûr, la nécessité de gérer l'apparition de clusters est légitime, mais elle ne peut se traduire par le maintien de prérogatives très exorbitantes du droit commun, qui autoriseraient le Premier ministre à restreindre les libertés sur des parties importantes du territoire.

nous ne pouvons admettre la suppression de l'article 1 A, que le Sénat avait introduit en première lecture. Cela revient à maintenir entre les mains du ministre de la santé des prérogatives larges et indéfinies pour lutter contre l'épidémie, sans garanties pour nos concitoyens. La fragilité juridique de ce régime a justifié, il y a quatre mois, l'instauration d'un régime d'exception, afin de sécuriser l'action des pouvoirs publics et d'encadrer les atteintes portées aux libertés. Il serait pour